Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Action extérieure de l'État » sont stables en valeur en 2020, à hauteur de 2,9 milliards d'euros. Cette stabilité apparente masque en réalité une augmentation des crédits de paiement de 1,1 % à périmètre constant, puisque le programme consacré à la présidence française du G7 prend fin le 31 décembre 2019.

quelques variations significatives de crédits devraient néanmoins caractériser l'année 2020. Les évolutions à la hausse correspondent essentiellement à l'augmentation de 24,6 millions d'euros de la subvention de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE),

À l'inverse, les évolutions à la baisse correspondent à une économie de constatation de 7,6 millions d'euros sur les contributions internationales, essentiellement liée au repli des contributions en faveur des opérations de maintien de la paix, une diminution de 8 millions d'euros des dépenses de protocole et à la baisse d'un certain nombre de subventions allouées aux opérateurs : Atout France, alliances françaises, Institut français de Paris.

L'effet change-prix sur les indemnités de résidence à l'étranger (IRE) et l'effet prix sur les rémunérations des agents de droit local (ADL) constituent les principaux facteurs d'évolution à la hausse de la masse salariale. Par ailleurs, l'effet du glissement vieillesse-technicité (GVT) sur la masse salariale de la mission est positif en 2019 et beaucoup plus important que les années précédentes. Il s'élève à près de 9 millions d'euros. Pour la première fois depuis 2012, la part du GVT qui correspond au remplacement d'agents ayant une certaine ancienneté par des agents plus jeunes, qui est habituellement négative, est positive. Le Gouvernement m'a indiqué que cette situation était notamment liée à la requalification des agents de droit local sur des postes plus qualifiés. J'avoue être un peu surpris que les agents de droit local puissent avoir un effet sur le GVT.

Troisièmement, le PLF 2020 prévoit pour la première fois un mécanisme de provision des effets de change-prix sur la masse salariale. Cela devrait permettre de limiter la surexécution chronique des dépenses de personnels

Nous souhaitons appeler l'attention sur le risque d'impasse du budget de l'immobilier à l'étranger. La chute importante des produits de cessions, qui traduit notamment l'épuisement du volume de ventes potentielles, fait peser un risque important sur le budget de la mission « Action extérieure de l'État

incompréhension entre Bercy et le ministère des affaires étrangères. Le travail doit se poursuivre. Nous avons l'impression d'un décalage entre les indemnités de résidence à l'étranger qui sont versées et les indemnités de résidence à l'étranger théoriques telles

d'août dernier, lors de la conférence des ambassadeurs, vous avez réaffirmé l'ambition de la politique d'influence de la France, que vous décrivez comme « l'un des trois piliers fondamentaux de notre politique étrangère globale La hausse des crédits du programme 185, « Diplomatie culturelle et d'influence », de près de 3 % par rapport à l'an dernier, semble témoigner de cette priorité politique.

Après une baisse des crédits en 2017 et une stabilisation l'an dernier, cette hausse est évidemment une bonne nouvelle et, pour beaucoup, un soulagement. Elle permet d'aller vers l'objectif, fixé par le Président de la République, de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans son réseau d'ici à 2030, sans néanmoins- je tiens à le souligner -être suffisante pour l'atteindre. Si les éléments que je viens d'évoquer pour l'enseignement français à l'étranger sont positifs, on ne peut pas en dire autant s'agissant des trois autres opérateurs du programme : Atout France, Campus France et l'Institut français. Ainsi, la subvention pour charge de service public accordée à Campus France est maintenue à son niveau de l'an dernier, soit 3,8 millions d'euros. Mais cet opérateur est chargé de mettre en oeuvre l'objectif présenté par le Premier ministre l'an dernier dans la stratégie d'attractivité universitaire « Bienvenue en France », qui vise à accueillir 500 000 étudiants étrangers en France de pays d'origine plus diversifiée qu'actuellement C'est aussi dans ce cadre que des frais de scolarité différenciés ont été mis en place, avec les contestations que nous connaissons dans le monde universitaire. Ces dernières ont poussé le Premier ministre à annoncer le triplement des bourses d'études et de stages, ainsi que certaines exonérations des droits d'inscriptions. Comment l'opérateur Campus France pourra-t-il faire face à ces nouvelles mesures sans augmentation de sa subvention ? Comment justifier le maintien du niveau des bourses dédiées aux étudiants étrangers au même niveau que l'an dernier dans ce contexte ? Pour répondre à ces interrogations, nous souhaiterions d'ailleurs qu'un bilan détaillé de l'utilisation de l'enveloppe dédiée aux bourses puisse être établi à l'occasion de la prochaine loi de règlement.

La subvention à l'Institut français, dont je veux saluer la qualité du travail, retrouve cette année son niveau de 2018, après une hausse de 2 millions d'euros l'an dernier. d'euros l'an dernier. Celle-ci était alors justifiée par la mise en oeuvre du plan pour la langue française et le plurilinguisme annoncé par le Président de la République.

Redéfinir notre politique d'attractivité touristique, mutualiser les moyens avec Business France, revoir le rôle de chacun des acteurs de cette politique ... pourquoi pas ? Mais Atout France a aussi besoin d'une visibilité pluriannuelle sur les crédits qui lui seront accordés pour réaliser ces économies dans les meilleures conditions. Cette visibilité doit lui être donnée dans le cadre de son nouveau contrat d'objectifs et de moyens. Nous y serons attentifs.

Près de 2 millions d'euros sont consacrés à ces réformes, qui reposent notamment sur la mise en place du vote par internet, l'élargissement des horaires, l'état civil électronique et la création d'une plateforme téléphonique d'accueil consulaire. Cette Cette modernisation de l'administration consulaire est évidemment souhaitable, mais elle est parfois difficile tant pour les agents dans les consulats et les ambassades que pour les Français de l'étranger. Alors que la demande de présence de l'État est toujours plus forte pour nos concitoyens à l'étranger, l'existence d'un lien humain demeure- nous le savons -fondamentale, et le numérique ne peut pas toujours le remplacer.

ont besoin d'un accompagnement important pour faire face à ces changements d'ampleur, dont les gains de productivité ne sont d'ailleurs pas toujours assurés et devront être vérifiés.

mission « Action extérieure de l'État », qui est pourtant le plus petit des budgets régaliens de la République, a déjà grandement contribué aux efforts de maîtrise des dépenses publiques depuis une quinzaine d'années.

En 2020 se poursuivra la réorganisation des modes de gestion des réseaux de l'État à l'étranger. Mais tous les ministères ne jouent pas le jeu et n'acceptent pas que l'ambassadeur devienne le pilote de l'ensemble des réseaux de l'État à l'étranger. C'est pourtant légitime et indispensable. Nous en reparlerons lors de l'examen du projet de loi d'orientation sur l'aide au développement, car la question se posera s'agissant de l'aide publique au développement. J'en viens maintenant au modèle de gestion immobilière du Quai d'Orsay. Il n'est pas soutenable, car il fait dépendre l'entretien courant des bâtiments des recettes exceptionnelles des cessions d'immeubles à l'étranger. l'étranger. Nous arrivons à une impasse dans ce domaine : l'État s'appauvrit et les possibilités de vente diminuent ! « Les prévisions de recettes sont inférieures à 30 millions d'euros. On a même plafonné à 4 millions d'euros en 2019, alors que le besoin réel est compris entre 40 millions d'euros et 80 millions d'euros par an. Il faut mettre un terme à l'érosion du patrimoine qui découle de cette gestion non vertueuse. La commission demande aussi au Gouvernement de réfléchir au projet de rénovation du Quai d'Orsay, dit QO21. « Mal adapté aux besoins, avec des espaces sans lumière, de lieu de restauration du personnel, ce projet est au point mort depuis un an, accumulant retard et dépassement du budget, qui atteint déjà 95 millions d'euros, pour moitié financés par des cessions de biens immobiliers à l'étranger. Pourquoi ne pas profiter de ce blocage au stade de l'avant-projet sommaire pour redéfinir le projet ? Celui-ci ne doit pas être un totem. » La parole est

Un effort est fait, et une provision de 15 millions d'euros est prévue. Plus globalement, les effets de change et l'inflation posent un problème de soutenabilité au programme 105. Nous devons donc être vigilants et veiller à ce que cette provision compensant les effets change-prix soit désormais annuelle. De même- là encore, c'est une demande récurrente de notre commission le Premier ministre a validé la couverture du risque d'une perte au change sur la rémunération des agents de droit local et sur les indemnités de résidence à l'étranger. Nous pouvons nous en féliciter. J'en viens à la sécurité des implantations diplomatiques, consulaires et culturelles. Les crédits budgétaires dédiés ont diminué en 2019, passant de 75 millions à 44 millions d'euros. Cette réduction a été compensée

La définition d'un programme d'investissements à la hauteur des besoins de financement et l'accroissement des dépenses éligibles au compte d'affectation sont nécessaires pour que cette réforme atteigne ses objectifs et que les crédits dédiés soient réellement consommés.

Nous avons émis un avis favorable sur les crédits de la diplomatie culturelle et d'influence, qui sont en légère augmentation du fait d'une hausse de 25 millions d'euros de la subvention à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). L'objectif énoncé par le Président de la République est de doubler les effectifs d'élèves scolarisés dans l'enseignement français à l'étranger d'ici à 2030, ce qui suscite plusieurs interrogations ; nous les avons évoquées en commission. « En premier lieu, on note une lente érosion de la part des enfants français scolarisés dans le réseau. Elle est passée en cinq ans de 38 % à 35 %. L'enveloppe des aides à la scolarité stagne et les droits d'inscription sont, eux, en constante augmentation. Le budget des aides à la scolarité suivra-t-il l'extension du réseau, donc du nombre de bénéficiaires potentiels ? Ou bien cette extension reposera-t-elle sur un modèle purement purement privé, dans une logique de " labellisation " des établissements, ce qui serait évidemment moins favorable ? « En deuxième lieu, on vise un doublement du nombre d'élèves, avec seulement 11 % de détachements supplémentaires

au fil de l'eau " ne permettrait pas de mettre en oeuvre les priorités du ministère des affaires étrangères ? Et ne risque-t-on pas de dénaturer le réseau en faisant reposer son extension sur un recrutement essentiellement local ? « En troisième lieu, le développement du réseau sur le plan immobilier est freiné par des obstacles à l'emprunt, qui doivent être levés. Ne faudrait-il pas alors autoriser l'AEFE à emprunter auprès d'établissements de crédit ? Elle ne peut le faire aujourd'hui. Un dispositif alternatif à l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger (Anefe) sera-t-il mis en place pour permettre le recours des établissements à la garantie de l'État ?

La France est aujourd'hui le cinquième pays d'accueil de ces étudiants. Elle est suivie de près par la Russie et le Canada. Plusieurs pays ont des stratégies très offensives. Je pense à la Turquie, dont le nombre d'étudiants internationaux a progressé de 180 % en cinq ans,

à de telles évolutions, notre stratégie d'attractivité est fragile. D'abord, les moyens qui lui sont consacrés sont insuffisants. Une politique d'exonérations a permis de limiter les effets de la hausse des droits d'inscription.

Par ailleurs, ces crédits ne sont pas intégralement consommés, ce qui est fâcheux. Cette année, seulement 76 % ont été effectivement confiés en gestion à Campus France. Plus généralement, comme l'a souligné la Cour des comptes dans un rapport récent, cette politique des bourses souffre d'un manque de stratégie d'ensemble. Elle doit être absolument mieux pilotée. Dans cette perspective, on pourrait envisager un rapprochement entre Campus France et Erasmus +, ce qui permettrait d'être plus efficace. Très bien ! Une meilleure articulation entre le réseau diplomatique et les établissements d'enseignement supérieur en France pour les étrangers est nécessaire. Les filières longues, les filières d'excellence, doivent évidemment être privilégiées sur les stages courts. Enfin, la politique des bourses doit être rendue plus visible sur le plan international par l'instauration d'une vraie marque, prestigieuse, avec une forte notoriété-

million d'euros, soit 0,6 %, alors que ceux qui sont destinés à la modernisation de l'administration consulaire sont en augmentation de 1,9 million d'euros. Ces deux chiffres illustrent la tendance de fond qui est à l'oeuvre dans le réseau consulaire depuis de nombreuses années, consistant à dégager des marges de manoeuvre grâce à la dématérialisation et la rationalisation rationalisation pour maintenir le service rendu aux usagers dans un contexte d'économies et de suppressions de postes. En 2020, les chantiers de modernisation vont se poursuivre, avec la mise en place d'un registre d'état civil électronique, le lancement d'un « centre mondial d'accueil consulaire » et le déploiement de l'application France-Visas, permettant un traitement entièrement dématérialisé des demandes de visas. Des marges de manoeuvre sont aussi recherchées dans des mesures de réorganisation. Il en est ainsi du regroupement d'activités, permettant des gains de productivité et des redéploiements d'effectifs. Dans les pays comptant plusieurs postes, des spécialisations sont mises en place, comme depuis le 1 septembre 2019 aux Émirats arabes unis : la compétence en matière de visas est exercée à Abou Dhabi, alors que celle en matière d'administration des Français est du ressort de Dubaï. Le projet de regrouper au service central de l'état civil à Nantes les transcriptions d'état civil, expérimenté depuis 2018 avec plusieurs postes en Europe, procède de la même logique et suscite quelques inquiétudes. Évoquons les réorganisations de la carte consulaire. Après la fermeture récente des consulats de Séville et de Moncton, après la transformation du consulat général de Boston en consulat d'influence, il est prévu en 2020 de supprimer un certain nombre de sections consulaires, notamment à Monaco et Tallinn, et de fusionner les fonctions de consul et de directeur de l'Institut français à Agadir, Bilbao, Fès et Tanger. Ces évolutions entament l'universalité du réseau. En 2020, comme depuis une décennie, l'administration consulaire continuera de se réformer pour maintenir le niveau de service rendu à une population de ressortissants français en augmentation continue de 81 % depuis 1998, et ce avec toujours moins de moyens. Afin de se conformer à l'objectif fixé par le plan stratégique Action publique 2022, prévoyant une réduction de 10 % de la masse salariale à l'étranger d'ici à 2022, le programme 151 supprimera encore 22 emplois en 2020, après 37 en 2019. Compte tenu des efforts de rationalisation déjà réalisés, comment ces suppressions de poste ne pourraient-elles pas se traduire, à terme, par une dégradation des prestations fournies ? Comment, dans ces conditions, préserver le contact humain avec le public, auquel les ressortissants français sont légitimement très attachés ?

Nos compatriotes, comme les quelque 3,5 autres millions de résidents étrangers installés au Royaume-Uni, devraient connaître une année particulière, celle du Brexit, aux conséquences aujourd'hui encore incertaines. raison pour laquelle nous nous sommes rendus à Londres. Nous avons pu échanger avec notre ambassadrice, le consul général et des membres de notre poste, dont je tiens à saluer à la fois l'engagement et le grand professionnalisme. présenter, monsieur le ministre, les principaux enseignements. D'abord, j'évoquerai le statut de résident pour les étrangers, qui doit leur permettre, après le Brexit, de vivre, de travailler, et d'étudier dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

Le premier concerne la vétusté de notre poste à Londres, qui impacte négativement les conditions d'accueil, d'une part, et de travail, d'autre part. J'y ajoute la nécessité de prendre, rapidement, les mesures de renforcement de la sécurité, s'agissant notamment des conditions d'accès. Le second point concerne plus largement la question des moyens dont dispose notre réseau pour assurer un service public de qualité, ce que j'évoquais au début de mon propos. Monsieur le ministre, les efforts demandés à votre ministère- 22 emplois supprimés en 2020 et 37 l'an dernier -ne sont ni tenables ni acceptables.

qui sont impactés par ces suppressions, que nous voterons contre les crédits de ce programme. Il s'agit d'une opposition utile au rayonnement et à l'action internationale de notre pays. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits destinés à notre diplomatie culturelle et d'influence augmentent en 2020. Je salue cet effort budgétaire, qui rompt avec la baisse drastique ayant prévalu sous le précédent quinquennat. Derrière cette progression globale du budget se cachent toutefois des disparités dans le traitement réservé aux opérateurs de notre diplomatie culturelle. et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Le relèvement de sa subvention était très attendu depuis la coupe franche qui avait fortement ébranlé le réseau en 2017. Ces moyens supplémentaires constituent donc une bonne nouvelle pour l'AEFE. deux bémols s'agissant de la politique d'expansion du réseau. Le choix de faciliter l'homologation de nouveaux établissements n'est pas sans soulever des inquiétudes sur le maintien d'un haut niveau de qualité de l'enseignement. En aucun cas, l'excellence de notre réseau ne doit être sacrifiée sur l'autel de son élargissement. En outre, il ne faudrait pas qu'une moindre attention soit portée à la situation, parfois délicate, des anciens établissements. Un juste équilibre doit donc être trouvé entre essor du réseau et soutien aux structures existantes. Sur l'ambition présidentielle de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'ici à 2030, je reste dubitatif sur le niveau des moyens qui permettraient de la concrétiser. J'en viens à la nouvelle stratégie pour l'accueil des étudiants étrangers : Bienvenue en France. Étonnamment, elle ne donne pas lieu à une augmentation de la subvention versée à son opérateur, Campus France. La stabilisation de son montant n'est assurément pas à la hauteur de l'objectif de 500 000 étudiants étrangers accueillis d'ici à 2027. Le contexte concurrentiel international imposerait d'avoir enfin les moyens de nos ambitions. Je tiens également à alerter sur l'utilisation des crédits destinés aux bourses versées aux étudiants étrangers. J'ai appris qu'ils ne leur sont, depuis 2016, pas entièrement consacrés. du delta, le ministère n'est pas en mesure de nous dire précisément ce qu'il en est ... C'est inquiétant ! Le troisième opérateur de notre diplomatie d'influence, l'Institut français, ne bénéficie pas d'un traitement favorable en 2020. Après le coup de pouce de l'année dernière, sa subvention retrouve son niveau de 2018, et je n'évoquerai même pas l'état déplorable des bâtiments, notamment à Mexico. Il s'agit clairement d'un repli par rapport aux ambitions du plan Langue française et plurilinguisme, dont certaines actions ne pourront sans doute pas être déployées. Quant au rapprochement de l'Institut français avec la Fondation Alliance française, si la procédure a bien avancé sur le plan fonctionnel, elle est bloquée sur le plan matériel. Je m'étonne que le ministère se refuse à jouer les arbitres sur ce point. Au final, je porte sur ce budget une appréciation en demi-teinte l'indéniable hausse des crédits permettra de valoriser notre réseau d'enseignement français à l'étranger, mais elle exerce en quelque sorte un effet d'éviction sur les autres piliers de notre politique d'influence. Aussi, au regard des réserves soulevées,

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la voix de la France est écoutée dans le monde et elle doit continuer de l'être. La situation internationale n'est pas sur le chemin de la stabilisation. C'est peut-être encore moins le cas depuis que les alliances sont devenues changeantes et que les accords sont susceptibles d'être remis en cause à tout moment. La diplomatie est cependant un outil essentiel dans la politique internationale. Son action se fait souvent dans l'ombre. Ses échecs sont davantage remarqués puisqu'ils se traduisent trop souvent par des guerres. La diplomatie évite parfois les conflits, mais elle participe surtout à bâtir ou rebâtir la paix. À cet égard, la France doit maintenir des capacités diplomatiques de haut niveau pour continuer de faire rayonner ses idées et ses valeurs. Ces capacités nous permettent également de connaître en détail nos interlocuteurs, ainsi que les situations et les enjeux auxquels il nous faut faire face. L'année dernière, le réseau diplomatique français a reculé de la deuxième à la troisième place, derrière les États-Unis et la Chine. Il nous faut impérativement maintenir notre rang si nous souhaitons que notre pays reste une grande puissance de diplomatie et de paix. France poursuit son effort et nous nous félicitons que les budgets du ministère de l'Europe et des affaires étrangères soient en hausse. Les crédits de la mission « Action extérieure de l'État » sont, quant à eux, maintenus. Afin de procéder aux économies nécessaires, l'État s'est lancé dans une réforme visant à rationaliser les moyens dont il dispose à l'étranger. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'est engagé avec rigueur et sincérité dans la mutualisation des moyens de l'État à l'étranger, ce qui est à saluer. La logique de cette réforme nous semble être la bonne, et nous souhaitons la voir aboutir. Plus généralement, nous nous interrogeons sur les moyens de parvenir aux objectifs que souhaite atteindre le Gouvernement. Il nous semble que des pistes d'amélioration subsistent. Le nombre d'équivalents temps plein baisse en dix ans de presque 10 % et, sur la même période, les dépenses de personnel ont augmenté de 34,5 %. Même si l'inflation explique en partie ce phénomène, cette tendance nous semble problématique. Nous sommes plusieurs à déplorer la baisse des effectifs, mais nous sommes encore plus nombreux, me semble-t-il, à regretter que cela se traduise tout de même par l'augmentation des dépenses de personnel. De même, le produit des ventes immobilières est en forte baisse. C'est inquiétant parce que cela signifie qu'il n'y a plus beaucoup de « bijoux de famille » à vendre ! Vous nous avez dit, monsieur le ministre, être conscient que « nous ne pouvons pas vendre que « nous ne pouvons pas vendre indéfiniment nos emprises majeures à l'étranger ». Il s'agit à présent de s'orienter vers la recherche de sources d'économies durables. Vous nous avez rassurés sur le devenir de la diplomatie culturelle et d'influence, qui est, comme vous avez eu l'occasion de le rappeler, une diplomatie stratégique. Nous nous réjouissons que vous ayez stoppé la diminution des crédits qui y sont affectés et recommencé à les faire augmenter. Cette diplomatie est essentielle, car elle donne du poids aux prises de position de la France. Elle promeut nos valeurs et notre modèle. Le pays des droits de l'homme doit avoir une voix qui porte. Plus la France enseignera aux étrangers, plus la France sera écoutée. Il faut donc saluer l'objectif de doublement des effectifs des écoles françaises à l'étranger à l'horizon 2030. Nous entendons les inquiétudes sur l'existence des financements permettant d'atteindre cet objectif. Nous souhaitons vous voir réussir : il faudra donc que les moyens nécessaires soient mis en oeuvre pour y parvenir. Nous savons que l'enseignement aux étrangers est crucial, et nous sommes confortés dans cette idée lorsque nous regardons nos voisins. Plusieurs pays se sont effectivement engagés dans une démarche d'influence l'enseignement à l'étranger ou aux étrangers. C'est ainsi que le nombre d'étudiants étrangers en Turquie a augmenté de 180 % ces % ces cinq dernières années. Nous ne devons pas relâcher nos efforts. Il a été fait état de difficultés dans l'obtention de visas français par les étudiants étrangers. Il nous semble qu'une clarification des procédures et une accélération du traitement des dossiers soient nécessaires. La stratégie diplomatique française ne doit pas être mise à mal par des problèmes d'organisation des services : les visas doivent être délivrés en temps utile. Sur tous les sujets qui ont trait à son action extérieure, la France doit maintenir son effort. Nous sommes moteurs en Europe et nous sommes force de propositions sur la scène internationale. Cette dynamique doit être conservée et amplifiée. Les années à venir s'annoncent porteuses de tensions et de dissensions. L'échange et la négociation sont les alternatives à l'emploi de la force. Nous qui n'oublions pas le prix du sang savons qu'il faut donner les meilleures chances à la diplomatie si nous voulons maintenir la paix. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous évoluons dans un monde en pleine recomposition géopolitique et stratégique, dans lequel les anciennes puissances sont concurrencées par de nouvelles, la Chine et l'Inde, des puissances d'abord économiques mais désormais politiques, qui souhaitent aussi peser sur l'ordre du monde. Cet ordre du monde est, hélas, loin d'être en ordre. De nouveaux défis se présentent : le changement climatique et ses probables effets en termes de migrations, ou encore l'expansion du numérique, qui, si elle n'est pas encadrée, peut être une source de dérives. Toujours, des conflits perdurent et d'autres éclatent. Au-delà du Proche-Orient, je pense aussi au continent sud-américain, dont plusieurs pays sont en proie à des difficultés politiques : le Venezuela en particulier avec l'intransigeance de son dirigeant, mais aussi l'Équateur, la Bolivie, le Chili et la Colombie, dans lesquels les contestations s'étendent. Aussi, dans ce contexte, la France doit absolument tenir sa place pour défendre la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Comme l'a rappelé le Président de la République lors de la dernière conférence des ambassadeurs, « l'esprit français, c'est un esprit de résistance et une vocation à l'universel ». Refuser la fatalité, diffuser l'humanisme qui nous est cher impliquent pour la France de conserver son rayonnement sur la scène internationale. La mission « Action extérieure de l'État » que nous examinons aujourd'hui est le levier de cette ambition. Elle n'est pas la seule. La politique d'aide au développement et la politique du ministère des armées l'accompagnent à bien des égards. S'agissant de la défense, je n'oublierai pas de saluer la mémoire des treize militaires exceptionnels qui, au Mali, ont payé de leur vie leur engagement au service de la paix dans le monde. Mes chers collègues, comme l'a exposé le rapporteur, les crédits de la mission sont stables en valeur et conformes à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. On peut toutefois observer que la fin du programme consacré au G7 entraîne en réalité une hausse de 1,1 % des crédits de paiement. J'en profiterai pour rappeler que le G7, qui s'est déroulé à Biarritz, a démontré que l'efficacité diplomatique pouvait être encore au rendez-vous malgré la crise du multilatéralisme. Pays organisateur, la France s'est retrouvée au coeur d'annonces importantes parmi lesquelles la reconstitution du Fonds vert pour le climat ou la réaffirmation de l'Afrique comme zone prioritaire de l'aide au développement. Dans le détail de ce budget, je partagerai les observations de la commission, en particulier sur la question de la chute importante des produits de cessions qui menace le budget de l'immobilier à l'étranger, la pression qui pèse sur certains opérateurs auxquels on demande de participer à l'effort de rationalisation des moyens dans le cadre d'Action publique 2022, ou encore les conséquences que pourrait avoir sur le lien entre les Français de l'étranger et leurs services publics une modernisation à marche forcée de l'administration consulaire. On peut en revanche se féliciter du renforcement, à hauteur de 24,6 millions d'euros, du budget de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dont la subvention pour charge publique avait tout de même diminué de 33 millions d'euros en 2017. On le voit, nous revenons de loin ! Cet abondement est plus que nécessaire pour remplir l'objectif, décidé par le Président de la République, de doubler le nombre d'élèves scolarisés au sein du réseau français. Disons-le, la francophonie est en perte de vitesse. Aussi, il apparaît essentiel de préserver les moyens des quelque 522 établissements français qui accueillent 200 000 élèves étrangers sur un effectif total de 365 000. Il faut bien mesurer l'enjeu de la diffusion de notre langue. Encourager au maintien du plus grand nombre possible de locuteurs français, c'est conserver un levier fort de la transmission de nos valeurs, dont le caractère universel est encore-on s'en réjouit ! -reconnu dans le monde. Enseigner le français, c'est en quelque sorte enseigner la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est vrai ! La coopération culturelle passe aussi par le développement et le renforcement d'une approche partenariale. Le nouveau traité d'Aix-la-Chapelle, signé en janvier dernier avec l'Allemagne, élargit et renouvelle le champ de la coopération culturelle entre Berlin et Paris. J'en suis heureux et j'espère que les projets communs, que ce soient la plateforme numérique et les instituts franco-allemands intégrés contribueront à valoriser la relation franco-allemande, dont on connaît tous l'impact politique sur la scène internationale. Enfin, c'est bien sûr au travers de la conservation d'un réseau dense dense d'ambassades que la France exerce son rayonnement. À mon sens, le réseau diplomatique doit conserver, autant que faire se peut, son universalité. Pour autant, c'est un objectif qui n'interdit pas un redéploiement plus net des moyens d'un poste diplomatique à un autre, en particulier pour répondre au souhait du chef de l'État de voir la France exercer davantage son rôle de puissance d'équilibre dans certaines régions du monde, en Asie par exemple. À cet égard, la volonté de construire un partenariat euro-chinois du XXI siècle est à mettre en oeuvre. Mes chers collègues, dans cette perspective d'approfondissement de l'action extérieure de l'État dans le monde, le RDSE soutiendra les crédits ouverts

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'an dernier, le Président de la République a annoncé vouloir doubler le nombre d'apprenants du français, alors même que les prédictions démographiques anticipent un milliard de locuteurs d'ici à 2065. L'AEFE a donc intégré 8 800 nouveaux élèves et labellisé 30 nouveaux établissements. Toutefois, le détachement de nouveaux enseignants et l'augmentation de la subvention de 25 millions d'euros seront difficilement suffisants pour absorber le choc.

Bref, la plupart des outils censés viser un double objectif de rayonnement culturel et de développement de la francophonie doivent toujours faire plus, avec moins. Je souhaiterais aborder ici le plan Bienvenue en France. Même en modifiant les règles de calcul avant l'été, certaines zones d'origine prioritaires, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne entre autres, avaient vu le nombre de demandes baisser de 24 % et 14 %. Monsieur le ministre, quelle sera votre action à ce sujet après la décision historique du Conseil constitutionnel du 11 octobre dernier rappelant le nécessaire respect des exigences de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction ? L'autre levier essentiel de notre diplomatie, c'est bien évidemment le réseau administratif et politique auprès de nos compatriotes à l'étranger et des étrangers souhaitant avoir des liens avec la France. Certes, l'objectif fixé dans le cadre de CAP22 d'une réduction de 10 % des effectifs a été ramené à 5,7 %. Mais il faut quand même rappeler que le personnel diplomatique a baissé de 9,4 % depuis quinze ans. Pour 2020, ce sont 81 postes qui sont supprimés sur la mission. Mes chers collègues, la précarisation de notre réseau consulaire est préoccupante. L'an dernier, plus de 150 demandes de missions de renfort n'ont pu être satisfaites par les services du ministère, faute de personnel. En parallèle, on estime que le cumul des congés non pris et des heures non rémunérées et non récupérables équivaut à 70 emplois à temps plein. La situation est similaire à celle de l'année dernière. S'il faut s'interroger, comme l'ont fait nos collègues Rémi Féraud et Vincent Delahaye sur l'augmentation de la charge de l'indemnité de résidence à l'étranger, me semble-t-il, avec une extrême prudence. En effet, certaines villes du globe deviennent si chères que l'indemnité se révèle parfois nettement insuffisante pour vivre dans de bonnes conditions.

coûte beaucoup plus cher que le recrutement de fonctionnaires. Mon groupe constate une grande différence entre les attentes et les moyens mobilisés, et ce encore plus au regard des priorités fixées par le Gouvernement, que je rappelle : l'action pour la paix et la stabilité, la promotion de l'Union européenne, la défense de la démocratie et des droits humains, et, enfin, la régulation économique et commerciale.

Les choix diplomatiques de notre pays s'appuient de plus en plus souvent sur des considérations d'alliance et/ou économiques, plutôt que sur des analyses de la situation. Nous avons le sentiment que notre réseau et ses personnels sont- pardonnez-moi ce terme ! -des « VRP » des produits français, notamment, et surtout, en matière de commerce des armes. Vous connaissez notre opposition sur ce sujet. Comment poursuivre un objectif de promotion de la paix tout en étant l'un des plus grands exportateurs d'armes ? Vous l'aurez compris, mes chers collègues,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai par le programme 105 de la mission « Action extérieure de l'État », relatif aux ambassades et à l'action diplomatique. Il prévoit une légère hausse du montant global des crédits, qui s'élèvent à 1,78 milliard d'euros pour 2020. Premier point notable : la très légère diminution des contributions obligatoires de la France, qui représentent 676 millions d'euros. J'ai fait partie de la délégation de notre commission qui était à l'ONU en début de semaine. Je souhaite saluer notre équipe diplomatique, conduite par Nicolas de Rivière. La France est le cinquième ou sixième contributeur à l'ONU. Notre rang de membre permanent du Conseil de sécurité nous y oblige et nous devons souscrire à des contributions obligatoires. Mais si nous regardons les contributions volontaires, avec 45 millions d'euros, notre contribution est faible et nous ne pointons qu'à la quinzième ou vingtième place. Il faut être attentif à cette situation, car un déclassement dans ce domaine entraîne une perte d'influence. Le deuxième poste de dépenses du programme 105 est consacré au fonctionnement du réseau diplomatique à l'étranger, soit 621,6 millions d'euros. J'appuie votre choix de proposer une légère progression pour ce poste. Nous soutenons votre réforme consistant à mutualiser et à moderniser les services de l'État français à l'étranger. Mais la réduction des crédits recherchée ne doit pas altérer la bonne exécution des missions. Ce n'est pas le cas ! Ce qui nous inquiète dans ce programme 105, c'est la politique immobilière du Quai d'Orsay. L'image que donne notre diplomatie est celle d'un reflux continu depuis 1995. Pour financer l'entretien de notre patrimoine, nous cédons des propriétés parfois emblématiques. J'ai arrêté ! Vendre les « bijoux de famille » pour financer son train de vie a une fin. Et nous y sommes

Déjà l'an dernier, je vous indiquais qu'il fallait penser différemment sur le sujet. En commission, vous nous avez demandé de faire des propositions. En voici : à Addis-Abeba, par exemple, notre ambassadeur serait en mesure de réaliser ses propres recettes pour entretenir sa résidence et ses trente-sept hectares de végétation, le tout sans puiser dans les deniers publics. Pour y parvenir, il faut réformer la comptabilité publique pour donner de l'autonomie à nos chefs de poste, afin de leur permettre de gérer au mieux localement notre patrimoine sans nécessairement faire appel aux deniers publics. du programme 151, qui concerne les consulats et les Français de l'étranger- dont je fais partie -, nous devons faire face à une situation où nous avons de plus en plus d'expatriés ou de personnes de passage, mais de moins en moins de moyens : c'est le fameux effet ciseau. J'approuve les mesures d'adaptation que vous avez prises dans ce domaine. Mais cela ne suffira pas à dynamiser le réseau consulaire, constitué de 206 postes et d'un réseau d'environ 500 consuls honoraires, que je salue, car leur action bénévole est essentielle à son bon fonctionnement. Là encore, notre réseau consulaire donne l'image d'un repli permanent : la fermeture des consulats de Moncton et de Séville, la transformation du consulat général de Boston en consulat d'influence, etc. J'arrête là Quelle sera la carte consulaire dans dix ans ? Voilà la question ! Ce réseau doit être abordé non pas comme une structure de coûts, mais comme une opportunité de gérer des revenus. Si l'intégralité des recettes des visas était affectée à ce programme 151, notre présence consulaire pourrait ainsi s'étendre hors de nos frontières sans que cela coûte un sou au contribuable. On pourrait aussi s'inspirer des bonnes pratiques les consuls honoraires allemands peuvent effectuer les prises d'empreintes biométriques, ce qui évite aux Allemands de faire de longs déplacements pour pouvoir renouveler leurs passeports. De plus, cela nous permettrait de faire des économies de fonctionnement substantielles. du programme 185, qui concerne notre diplomatie culturelle, je soutiens sans réserve la dynamique initiée par le Président de la République dans le but de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans l'enseignement français à l'étranger à l'horizon 2030. Pour y parvenir, vous avez présenté une réforme de l'enseignement français à l'étranger. Afin de soutenir le développement du réseau, vous avez augmenté la subvention de l'AEFE de 24,6 millions d'euros. Mais Bercy veille : avec une augmentation de la réserve de précaution de 3 % à 4 % du budget de l'AEFE, la dotation de l'État ne représentera en fait que 16,15 millions d'euros. Mon collègue Jean-Marie Mizzon reviendra plus en détail sur ce programme 185, tout comme j'y reviendrai au cours des débats. Puisqu'il me reste quelques secondes, je veux rendre hommage, monsieur le ministre, à votre action personnelle à la tête de ce ministère : je n'entends que des éloges à votre égard. Je voulais le signaler. La parole

Votre constat était très clair : « Les grandes puissances sont résolues à faire de l'Europe leur terrain de jeu. [ ...] Le système multilatéral est la cible d'attaques sans précédent. [ ...] La grande compétition mondiale [ ...] se joue sur des terrains nouveaux. Notre commission partage votre analyse. Quand on regarde le monde avec lucidité, comme vous nous invitez à le faire, il y a de quoi être saisi de vertige. une aggravation accélérée des menaces : menaces de la force, comme on le voit dans le nord-est Syrien, mais aussi en mer de Chine, et jusqu'en Méditerranée, dans les eaux territoriales d'un État membre de l'Union européenne ; menaces de la faiblesse, celle des États faillis, terreau du terrorisme djihadiste, comme notre pays ne le sait que trop au Sahel. Je rends à cet instant un nouvel hommage à l'action résolue et courageuse de nos armées et je salue la mémoire de nos treize militaires morts au combat, morts pour la France, au Mali.

nouveaux espaces de conflictualité : après le cyberespace, l'espace extra-atmosphérique, pour lequel la France et l'Europe doivent rester des acteurs de premier plan. Je me félicite à cet égard de l'ambition portée par le conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne de Séville, qui a prévu un engagement financier très fort, lequel fera de l'Europe un acteur de tout premier plan. Face à ces crises, les outils de régulation issus de la Seconde Guerre mondiale sont malheureusement contestés : le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué sur la Syrie, sur le Yémen, sur le conflit israélo-palestinien.

Le droit international est bafoué, la liberté de circulation des mers est contestée, les traités de maîtrise de la prolifération chimique et nucléaire sont fragilisés. Après la dénonciation du traité sur l'armement nucléaire intermédiaire, le traité FNI, c'est désormais le traité New Start de réduction des armes nucléaires stratégiques qui est en danger. En vérité, c'est tout le système de maîtrise de la prolifération nucléaire en Europe qui est menacé ! Sur notre sol ! Qui aurait cru cela possible il y a seulement quelques années ? On pourrait ajouter le retrait américain de l'accord nucléaire iranien, la stratégie dite de la « pression maximale », qui achève de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang sans régler aucune des trois principales menaces iraniennes : nucléaire, missiles balistiques, instabilité régionale. Même nos alliances les plus solides, comme la relation transatlantique, vacillent certains jours. L'opération turque dans le nord-est syrien a offert une victoire finale au régime de Damas et le retrait américain a livré aux Russes le Moyen-Orient. La menace djihadiste qui pèse sur l'Europe s'est hélas ! renforcée. Surtout, cela a montré que nos alliés américains pouvaient abandonner des alliés loyaux et efficaces- les Kurdes, et nous, la France, deuxièmes partenaires de la coalition -, et ce du jour au lendemain. Il n'est pas besoin d'avoir lu Clausewitz pour comprendre les conséquences désastreuses de l'offensive turque et de la complicité américaine sur les relations entre la Turquie, membre de l'OTAN, et les pays européens. Le

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, que j'ai l'honneur de présider, travaille à ce réveil stratégique européen en tissant inlassablement des relations étroites, tant en matière d'affaires extérieures que de défense, avec ses homologues des vingt-sept parlements de l'Union, Britanniques inclus. Le rapport sur la défense européenne de nos excellents collègues Ronan Le Gleut et Hélène Conway-Mouret, que je salue, a fait considérablement avancer la compréhension mutuelle. Nous n'hésitons pas à aller parler avec nos partenaires réputés les plus difficiles, nos collègues russes, avec lesquels nous allons entreprendre la rédaction d'un deuxième tome de ce rapport qui, à l'époque, avait marqué les esprits, ou les pays du groupe de Visegrad. Finalement, nous sommes surpris de l'écho rencontré, car ils ne sont, évidemment, ni aveugles ni sourds à l'évolution du monde Monsieur le ministre, la semaine prochaine, à Londres, seront fêtés les 70 ans de l'Alliance atlantique. Le secrétaire général de l'OTAN était hier à Paris. Il faut utiliser le moment de crise que nous vivons pour aller vers une Europe plus forte dans une OTAN plus forte.

de manière indépendante et crédible, car nous sommes dotés d'une armée disposant d'une autonomie stratégique fondée sur une capacité d'appréciation propre. La France n'a pas d'agenda caché ; elle ne vise qu'à produire de la sécurité et de la paix dans un monde devenu fou. Les rapporteurs de la commission, dans leurs rapports très fouillés, ont tous finalement posé la même question : celle du grand écart entre l'ambition et les moyens. Qu'il s'agisse des moyens des réseaux diplomatique et consulaire, optimisés jusqu'à l'extrême- pour le dire poliment -, ou du défi- le mot est -posé par l'objectif de doubler le nombre d'élèves apprenant le français d'ici à 2030, ce qui frappe c'est, bien sûr, le grand écart entre l'horizon des ambitions et, parfois, la petitesse des moyens mis à disposition pour l'atteindre. Nous savons- et je veux, ici, vous en rendre hommage et en porter témoignage -le combat que vous menez personnellement face à certains autres collègues ministres, situés sur la rive droite de la Seine, non loin du Val-de-Marne, pour tenter de maintenir et même d'accroître ces crédits. Je ne parle pas du modèle de financement des dépenses immobilières du Quai, notre bête noire depuis plusieurs années, car Ladislas Poniatowski l'a fait dans son rapport avec talent.

Nous attendons cela avec impatience. Malgré nos doutes, monsieur le ministre, nous soutenons votre action et celle de nos diplomates, auxquels je veux rendre hommage, engagés à vos côtés. La commission des affaires étrangères a donné un avis favorable à l'adoption de ces crédits, et j'espère que les réponses que vous nous apporterez nous conforteront dans nos choix. La parole est

Malheureusement, il continue à pâtir d'une image désuète, alors que les réformes qu'on lui impose depuis longtemps en font un ministère incroyablement moderne, dont le personnel montre une grande adaptabilité et une Vous allez vous opposer à nos amendements pour ne pas mettre en péril le subtil équilibre budgétaire validé par Matignon. Mais, franchement, ce ministère mérite mieux que les nouvelles économies qui lui sont imposées chaque année. Grâce à lui, la France a une place et une influence unique à l'étranger parce que nous figurons encore dans les trois premiers réseaux diplomatiques au monde. Mais, comme ses résultats sont plus qualitatifs que quantitatifs, et donc difficilement mesurables, il demeure la cible des coupes demandées par Bercy. Il est vrai que nos trois millions de compatriotes résidant à l'étranger n'ont aucun moyen de pression en dehors de la voix de leurs élus locaux ou au Parlement. Le constat de notre perte d'influence est partagé par tous. Alors, votre annonce d'un budget stabilisé ne changera rien à la triste réalité, tandis que notre présence à l'étranger décline parce que nous réduisons partout nos effectifs ou parce que nous disparaissons parfois en fermant nos missions, comme c'est le cas avec les consulats de Moncton ou de Séville. Monsieur le ministre, vous avez rappelé, lors de la conférence des ambassadeurs, l'objectif du Quai d'Orsay : « Faire preuve d'agilité, d'imagination, et, comme dirait le Président de la République, d'audace. » Mais à quelles fins ? Pour trouver comment continuer à faire la même chose avec des moyens financiers et humains toujours plus réduits ? Je puis vous assurer que nos diplomates font déjà preuve d'une incroyable créativité pour sauver la face et préserver l'image de notre pays, à commencer par l'organisation du 14-juillet. En fait, ce budget pour 2020 est un budget en trompe-l'oeil, même s'il paraît plus sincère que le précédent, puisque vous prenez en compte les effets de l'inflation mondiale sur les salaires et le risque d'une perte liée aux taux de change. Vous annoncez une dotation de 2,87 milliards d'euros, stabilisée, pour la mission « Action extérieure de l'État », avec même une légère augmentation de 2 millions Mais, au sein de cette enveloppe globale, de nombreux programmes sont en baisse. Par exemple, les crédits de l'action Réseau diplomatique baissent de 24 millions d'euros, ceux qui sont dédiés à la sécurité à l'étranger diminuent de 25 millions d'euros par rapport au PLF précédent. Les crédits du programme 105, « Action de la France en Europe et dans le monde » sont quasi stables, après, quand même, une baisse de 118 millions d'euros en 2018. Le plaisir suscité par la hausse de 3 % des crédits du programme 185 n'est qu'éphémère lorsque l'on constate, en même temps, la fermeture de quatre instituts français, dont celui d'Oslo, qui demeure pour moi incompréhensible. Pour être en contact avec nos élus de proximité, les conseillers consulaires, les personnels diplomatiques, éducatifs, culturels et économiques, je puis vous confirmer que plus aucune ambassade n'est épargnée par le manque d'investissement et de moyens humains. Il faut se déplacer sur le terrain pour voir des bâtiments trop souvent mal entretenus ou que nous sommes forcés de vendre, car nous sommes dans l'incapacité de les rénover ou parce que le produit de leur vente est attendu dans la contribution du ministère. Je crains fort que la rallonge de 8 millions d'euros que vous avez obtenue, monsieur le ministre, ne soit insuffisante pour l'entretien de notre parc immobilier.

d'ambassade (SGA) en sont un autre exemple, ces postes regroupant plusieurs fonctions sur une même personne. Ne poussons-nous pas la rationalisation à l'extrême, en fusionnant des métiers différents ? Le service public en pâtit, et nos compatriotes s'en plaignent régulièrement auprès des élus des Français de l'étranger ou à travers les sondages que nous faisons. L'image de la France s'en trouve également dégradée auprès des étrangers, pour lesquels le consulat est le premier contact avec notre pays. Monsieur le ministre, nous ne savons plus comment exprimer notre désarroi devant une situation que nous voyons se dégrader. Si nous étions à l'os il y a dix ans, où en sommes-nous aujourd'hui ? Allons-nous nous arrêter ? Eh bien, non ! Malgré l'artifice d'un budget stabilisé cette année, de nouvelles économies sont attendues sur la masse salariale, notamment avec la suppression de 81 équivalents temps plein. L'objectif est la diminution de 10 % de la masse salariale sur toutes les missions de notre réseau d'ici à 2022, soit la plus grande économie jamais imposée au Quai d'Orsay. Dans ces conditions, il est difficile d'envisager comment les services sur lesquels comptent les Français de l'étranger pourraient être améliorés. Ces économies se sont traduites par la suppression de 241 postes depuis deux ans. Derrière la froideur de ces chiffres, il y a des femmes et des hommes qui ont donné beaucoup au ministère, parfois pendant plusieurs décennies, en travaillant sous contrat local, et qui sont aujourd'hui licenciés.

La rationalisation des services dans le cadre de la réforme « Action publique 2022 » donne mission aux ambassadeurs de faire des propositions concernant notamment la mutualisation du personnel. C'est une excellente initiative, même s'il faut comprendre par mutualisation l'obligation de faire des propositions de suppressions de postes sur l'ensemble des services, et le ministère y a plutôt perdu, selon un rapport de l'Assemblée nationale.

l'influence française au-delà de nos frontières se mesure aussi par la préservation de notre rayonnement culturel, qui n'est pas épargné, puisque le PLF pour 2020 prévoit la baisse des subventions de tous les grands opérateurs, alors que votre gouvernement avait promis une hausse des crédits dédiés à la politique culturelle et d'influence. Or une économie de 1,2 million d'euros est réalisée sur le réseau des alliances françaises, du fait d'une diminution des crédits de sécurisation et d'un effort de rationalisation. Nous n'avons pas oublié la démission du de la Fondation Alliance française en janvier 2018,

Cet affaiblissement culturel semble bien entériné au sein de ce PLF, puisque France Médias Monde connaît une nouvelle baisse de ses crédits. TV5 Monde, qui avait déjà pâti l'an dernier de la non-répercussion de l'inflation, voit ses crédits simplement reconduits. Je vais maintenant passer à l'éducation et au budget de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, qui gère un vaste réseau, unique au monde, car les autres pays présents à l'international voient leur système éducatif soutenu par des établissements privés. Il n'est donc pas juste de comparer l'Agence aux établissements étrangers concurrents. Nous saluons la sanctuarisation des crédits de financement des aides à la scolarité, tant pour les élèves français du réseau des établissements de l'AEFE que pour les étudiants étrangers suivant leurs études en France. Nous sommes heureux de voir les moyens dévolus à l'Agence augmenter de 24,6 millions d'euros, mais cette hausse ne compense pas la suppression de 33 millions d'euros décidée en 2017. Il manque toujours 7 millions d'euros à la loi de finances pour 2019, D'autre part, cette coupe brutale de 2017 a entraîné la hausse des frais de scolarité liée à la participation forfaitaire accrue des établissements au budget de l'AEFE, qui est passée de 6 % à 9 %. Se pose alors la question de la prise en charge des demandes de bourses scolaires avec des frais plus élevés, dans une enveloppe financière maintenue à 105 millions d'euros. Enfin, le Président de la République a proposé de doubler le nombre d'élèves scolarisés d'ici à 2030, objectif téméraire, qui n'est basé sur aucune évaluation de la demande, mais que l'on ne peut qu'épouser, puisqu'il soutient la francophonie. A été annoncée dans la foulée la création de 1 000 postes d'enseignants titulaires supplémentaires sur dix ans, soit 100 postes par an pour répondre à la demande présidentielle. Mais, dans le même temps, vous lancez ce programme de recrutement par une baisse de 106 ETP en 2020 pour l'AEFE, monsieur le ministre. Rappelons que ce sont 512 postes qui auront été supprimés en trois ans. L'ambition est belle, et nous la soutenons volontiers, mais où sont les moyens ? Et comme il n'y a pas de petites économies, je vais ajouter à la liste la réduction de la dotation pour l'organisation en mai 2020 des élections consulaires, de l'ordre de 1,3 million d'euros. Vous avez affirmé que le nombre de bureaux de vote serait stabilisé ; certes, mais tel n'est pas le cas de celui des centres de vote, en forte diminution. Le vote électronique ne sera pas accessible à tous. Tout doit être fait pour que ces élections consulaires aient le taux de participation le plus élevé possible. Je puis vous assurer que ces élus sont devenus des relais indispensables de notre réseau diplomatique sous tension.

Nous ne pouvons pas voter ses crédits, qui ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, et nous ne voulons pas donner raison à Bercy, qui demande chaque année de nouvelles économies. Comprenez notre vote négatif comme un signe de solidarité envers les personnels, à qui l'on demande toujours plus sans leur donner les moyens, et comme une marque de soutien personnelle, monsieur le ministre, vous qui ne ménagez pas vos efforts pour défendre votre budget. La parole

décroissance des crédits et des effectifs. C'est un budget au service de la « diplomatie de l'audace » prônée par le Président de la République lors de la réunion des ambassadeurs.

me donne également l'occasion de saluer la mémoire de nos treize soldats tombés cette semaine au Mali. Pour ce qui concerne la masse salariale, le Gouvernement a pris la sage décision

J'en viens à présent à la diplomatie culturelle. Avec la hausse de la subvention allouée à l'AEFE, le plan de développement de l'enseignement français à l'étranger de ce dernier est cependant subordonnée à l'adoption d'une réforme des modalités d'octroi de la garantie de l'État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger. La situation est pour le moins paradoxale.

Je souhaite aussi connaître votre avis sur la proposition de la Cour des comptes consistant à confier à un seul opérateur le pilotage opérationnel de la mobilité internationale des étudiants, en d'autres termes le rapprochement

à propos de laquelle vous avez rappelé, monsieur le ministre, qu'elle était « l'un des trois piliers fondamentaux de notre politique étrangère globale ». La promotion de la langue française dans le monde et la valorisation du réseau d'enseignement français à l'étranger constituent à ce titre une composante majeure de notre diplomatie, et la commission de la culture y est bien entendu très attachée. En 2020, la subvention pour charges de service public de l'AEFE atteindra 408,6 millions d'euros, soit une augmentation de 24,6 millions d'euros ou de 6,4 %. Nous nous réjouissons de cette mesure, alors que l'annulation brutale de 33 millions d'euros au cours de l'été 2017 avait été très mal vécue par un réseau qui s'est senti fragilisé. Notre vigilance quant à la mise en oeuvre du plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, présenté en octobre dernier, sera donc à la hauteur de nos attentes le concernant. Un juste équilibre devra être trouvé entre le développement du réseau et le soutien aux structures existantes. Un autre grand plan est censé permettre à notre pays de rayonner à l'étranger, le plan Langue française et plurilinguisme. Alors qu'il est en grande partie piloté par l'Institut français de Paris, nous nous inquiétons du mauvais signal envoyé par la non-reconduction, certes annoncée,

Comme l'a indiqué son président lors de son audition, des arbitrages seront nécessaires entre les missions de l'organisme, du fait du manque de moyens. Ce plan, monsieur le ministre, est-il remis en question ? Au-delà de cette interrogation, nous nous réjouissons de la clarification des rôles entre les instituts français et les alliances françaises, grâce à la convention tripartite. Cependant, le rapprochement physique des deux opérateurs boulevard Raspail reste pour nous une vive source d'inquiétude. nous ne pouvons aborder la question de notre influence culturelle sans dire un mot de l'audiovisuel extérieur. La commission de la culture, en premier lieu sa présidente, ne cesse d'alerter sur la diminution constante de ses crédits, à rebours de nos ambitions.

Pour 2020, nous retiendrons que l'enveloppe globale de la mission atteint les 2,74 milliards d'euros. Cette stabilisation est en réalité directement liée à la disparition du programme relatif à la présidence française du G7. Je souhaite tout d'abord évoquer le contexte international, européen et ses impératifs. Cette séance est l'occasion de nous poser la question : « quel rayonnement et quelle influence voulons-nous pour la France ? », sachant que le rayonnement ne dépend pas que de l'état de notre réseau, sur lequel je vais évidemment revenir. En effet, rayonnement et attractivité sont liés. À quoi bon des capacités et des structures en nombre hors frontières si l'image et la situation intérieure de votre pays sont détériorées par de mauvais choix économiques, une recrudescence des violences, ou encore une crise sociale qui n'en finit plus ? La gestion des conflits sociaux résonne à l'international. Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités en la matière. Toutefois, ces fractures nationales, aussi importantes soient-elles, ne sauraient effacer l'importance de la singularité française sur la scène internationale, une singularité qui mérite d'être « réactivée » et « promue » ! La France ne peut rester spectatrice face à la fracturation accélérée de l'Union, écartelée par un Brexit interminable, déconnectée par les ultra-normes bruxelloises, déstabilisée par les vagues d'immigration et fragilisée par les différences de perception sécuritaire. Dans ce contexte international chahuté où les repères diplomatiques sautent, l'heure n'est plus au des années 2000. Nous sommes confrontés à une lutte d'influence exacerbée. Les domaines, le niveau d'excellence et les acteurs augmentent ! Les États-Unis, la Chine développent depuis près de quinze ans une stratégie offensive et inclusive. Les nouvelles routes de la soie sont loin d'être un simple concept. Il s'agit d'une nouvelle organisation globale, qui s'étend de Pékin à Djibouti, en passant par Gwadar. Je salue au passage les rapports de mon collègue Pascal Allizard sur ce sujet. Mais à ces géants du s'ajoute l'émergence de la Turquie, de l'Inde, de l'Arabie saoudite et de la Corée du Sud, qui consacrent à leur politique d'influence des moyens importants.

Elle a contribué à la démotivation et à la baisse des demandes. De fait, on assiste aujourd'hui à une sous-consommation des crédits. Cette ineptie résume bien une situation générale et révèle une certaine surenchère des réformes imposées au Quai d'Orsay. J'en viens à mon deuxième point, le réseau en lui-même. Les restructurations du réseau étaient destinées à mutualiser les moyens pour un meilleur accueil et une rationalisation des coûts. Cependant, après dix ans de réformes, le résultat dans certaines régions du globe est une rupture du lien de proximité entre les Français expatriés et leurs institutions. La volonté de maîtriser les finances publiques est bien évidemment primordiale, mais il semble que cette politique devienne contre-productive. Dans certains endroits où les prix des loyers sont très élevés, la vente du foncier s'est révélée être une erreur financière. Enfin, je veux vivement regretter l'insincérité de Bercy quant à l'utilisation du produit des cessions immobilières, qui devaient constituer des ressources exceptionnelles et bénéficier aux premiers acteurs de cette réforme, à savoir les agents.

Ils ont appelé à une refonte urgente de la gestion immobilière, et on ne peut que les soutenir. Concernant l'AEFE, ses crédits augmenteront de 24,6 millions. Nous souhaiterions saluer ce geste, si ces crédits n'étaient destinés à financer de nouvelles mesures, puisque le Président de la République s'est fixé comme objectif de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans les réseaux de l'enseignement français à l'étranger d'ici à 2030. Je me félicite de cette ambition, mais je m'interroge sur la réalité des moyens. Depuis 2013, ne pouvant emprunter sur des durées de plus de douze mois, l'AEFE bénéficiait d'avances de crédits provenant du compte de concours financiers. Cette année, ces avances ne sont pas reconduites, ce qui tend au respect de l'esprit de l'article 24 de la LOLF. Par ailleurs, l'Agence a commencé les remboursements à hauteur de 5,4 millions d'euros. Ces montages démontrent clairement que le financement de l'Agence n'est pas pérenne. Sans ces avances, l'AEFE se retrouve avec un défaut de trésorerie important, l'empêchant de financer des investissements, pourtant attendus, à Alger et à Moscou. Le montant évoqué est de 11 millions d'euros, ce qui laisse perplexe quant à l'augmentation de la somme allouée cette année. de l'étranger (Anefe) ? Grâce à cette association, 160 projets ont été garantis dans 110 établissements en quarante ans. La commission interministérielle d'octroi de la garantie de l'État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger vient d'être supprimée par décret. La suspension du dispositif empêche actuellement une quinzaine de projets d'être financés. Comment pouvez-vous justifier ces errements ? Enfin, je souhaite aborder un dernier point relatif à la représentation des Français de l'étranger. Depuis deux ans et demi, le Gouvernement et les députés de la majorité n'ont eu de cesse de revenir sur toutes les avancées que nous avions réussi à obtenir ces dernières années en faveur des Français de l'étranger. Le Sénat a adopté en janvier dernier, dans un large consensus, une proposition de loi visant à clarifier le droit électoral, reconnaissant aux élus de nouveaux droits. Cette proposition a été radicalement oubliée à l'Assemblée

Néanmoins, le rapporteur du projet de loi en a profité pour affirmer que les conseillers consulaires n'étaient pas élus, puis, reconnaissant son erreur, qu'ils n'étaient pas des élus comme les autres. Les conseillers consulaires du monde entier apprécieront ... Quand allez-vous donner aux conseillers consulaires les moyens d'exercer leur mandat ? Quand allez-vous leur donner de vrais pouvoirs, monsieur le ministre avons donc déposé une proposition de loi relative aux Français établis hors de France. Elle reprend le texte adopté par le Sénat, ainsi que tout ce que nos compatriotes demandent légitimement et que le Gouvernement leur refuse en matière fiscale et de droits sociaux. Cela dit, monsieur le ministre, nous voterons les crédits de cette mission, mais je ne peux que vivement vous inviter à prendre en compte les recommandations des rapporteurs pour l'avenir et à agir vite. L'expérience a démontré que la Haute Assemblée avait pour tort d'avoir raison trop tôt.

dans un monde instable, marqué par la multiplication des crises et la remise en cause des règles du jeu multilatéral, dans un monde en état d'urgence environnementale, certes riche en opportunités nouvelles, mais aussi en défis sans précédent, la France conduit une diplomatie à la fois audacieuse et pragmatique, pour défendre les intérêts de nos concitoyens, mais aussi les valeurs qui nous rassemblent.

trois chantiers nous occuperont de façon prioritaire. Le premier consiste à construire une véritable souveraineté européenne. Elle est indispensable si nous voulons avancer sur l'Europe de la défense, apporter une réponse commune au défi des migrations, accomplir un saut

Le deuxième chantier consiste à consolider le multilatéralisme renouvelé dont nous avons jeté les bases au cours de ces derniers mois, en lançant des coalitions d'action, notamment avec l'Allemagne, pour réunir les puissances de bonne volonté, sous la bannière sous la bannière de la coopération internationale, comme nous le faisons déjà dans l'Alliance pour le multilatéralisme. Le troisième chantier concerne ce que j'appelle les batailles nouvelles de l'influence. Dans le contexte d'une extension de la compétition internationale à tous les aspects de la vie culturelle et sociale, la culture,

l'ensemble de ces chantiers, nous avons besoin d'agir pour contribuer à la reconfiguration de l'ordre international que nous sommes en train de vivre,

Je veux d'abord rappeler que nous avons mis en oeuvre une première réforme : la réorganisation du mode de gestion des réseaux de l'État à l'étranger. Chacun a bien voulu, de manière quasiment unanime, reconnaître que cette réforme se mettait bien en place. bien en place. Aujourd'hui, les emplois de soutien et les crédits de fonctionnement de tous les réseaux internationaux de l'État sont effectivement sous la seule responsabilité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

c'est mon ministère qui est affectataire de l'ensemble du parc immobilier de l'État à l'étranger, ainsi que de l'ensemble des conventions de prestations que nous passons avec des partenaires locaux. Les crédits de fonctionnement servent à cela et, là aussi, nous avons eu les retours financiers nécessaires, à

reflète les montants que nous estimons nécessaires pour préserver le pouvoir d'achat des agents du ministère face à l'inflation. C'est une grande nouveauté et elle perdurera ! De la même manière, nous avons

à la gouvernance du nouvel ensemble et nous veillerons très attentivement à ce que la contribution à l'audiovisuel public soit répartie

bien ! Cette augmentation significative permet de répondre aux engagements qui ont été pris lors du discours du Président de la République à l'Académie française pour augmenter le nombre d'élèves

L'enjeu serait donc de représenter non plus la France, mais bien ses entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Cela nous laisse perplexes, notamment au regard du rôle des ambassades dans l'attribution et le fléchage de l'aide publique au développement. C'est pourquoi nous considérons qu'il est plus intéressant de renforcer les crédits de la diplomatie culturelle et éducative. De grandes ambitions sont portées par la francophonie, mais nos réseaux de diplomatie culturelle et d'enseignement ne disposent pas des moyens suffisants pour remplir leurs missions malgré un succès qui n'a jamais été aussi grand. Je voudrais évoquer l'exemple de l'université franco-tunisienne inaugurée cette année. Elle participe pleinement à cette image de structures réservées à une certaine élite. Comment Comment accepter la création d'un établissement, dont les frais d'inscription s'élèvent à 9 000 dinars, c'est-à-dire à peu près 2 900 euros, alors que le gouvernement tunisien a divisé par deux le budget des universités depuis 2008 ?

Conscient de l'impact de l'enseignement français à l'étranger, le Président de la République a souhaité que le nombre d'élèves scolarisés au sein du réseau double d'ici à 2030. Pour autant, dès la première année de ce gouvernement, l'AEFE a subi une annulation de crédits de 33 millions d'euros qui a entraîné la suppression de 512 postes sur trois ans.

Afin de compenser cette difficulté budgétaire et pour ne pas altérer la qualité des enseignements dispensés au sein du réseau, de nombreux établissements n'ont d'autre choix que d'augmenter les frais de scolarité. Ce sont par conséquent les familles, qui ne sont pas toutes aisées, contrairement à une idée reçue, qui souffrent le plus de cette baisse de subvention. Cet amendement vise à flécher 15 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires vers l'action n° 05, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au sein du programme « Diplomatie culturelle et d'influence » et à réduire de 15 millions d'euros les crédits de paiement de l'action n° 06, Soutien, au sein du programme « Action de la France en Europe et dans le monde

S'il y a moins de boursiers, tout va bien ; les familles peuvent payer les frais de scolarité. Il n'en est rien ! On constate que les bourses prennent en compte de moins en moins d'éléments et correspondent de moins en moins aux besoins des familles. Ainsi, dans certains établissements, la « part du fondateur » n'est pas prise en charge par les bourses scolaires.

nous nous sommes très fortement mobilisés pour l'école inclusive, laquelle nécessite aussi des accompagnements à l'étranger. Or très peu de ces aides sont aujourd'hui financées. Nous proposons donc qu'une bonne partie de cette augmentation des bourses soit utilisée

des agents accueillis sous le régime des recrutés locaux. On atteint les limites de cette pratique. En toute logique, les conséquences sont négatives tant pour les secrétaires généraux d'ambassade que pour les directions centrales et les agents. Pourtant, cette année encore, la baisse de 61 millions d'euros des crédits des affaires consulaires ne fait que confirmer cette dynamique de dégradation des conditions de travail de l'ensemble des fonctionnaires à l'étranger.

je suis tenté, sans perversité, mais avec un plaisir malin, de vous rappeler que la modification des règles d'attribution des bourses

tendait à montrer notre désaccord quant au manque de soutien financier et humain qui vous est apporté, monsieur le ministre. Il est étonnant que vous deviez vous battre de cette façon

la question de la sécurité, qui reste un motif d'inquiétude. Nos consulats ne sont pas simplement mobilisés contre les

On peut ainsi relever 2 millions d'euros en moins de dotation de fonctionnement aux établissements à autonomie financière, 2 millions d'euros en moins pour l'Institut français de Paris, 2 millions d'euros en moins pour Atout France et une réduction de 1 million d'euros pour les alliances françaises locales. Alors que le Président de la République a fait part d'objectifs ambitieux pour la promotion du français l'an dernier, on ne peut que constater la baisse des budgets de tous les opérateurs qui concourent au rayonnement de notre langue.

l'Institut français se trouve aujourd'hui en difficulté. Nous souhaitons donc relever de 7 millions d'euros les crédits de paiement de l'action Coopération culturelle et promotion du français, afin de doter les acteurs de moyens leur permettant de répondre aux ambitions affichées.

La décision de créer de nouveaux postes est prise lorsque des sujets d'actualité ou des problématiques prenant une ampleur particulière nécessitent qu'une personne soit clairement identifiée pour mener un plaidoyer spécifique. Le nombre de ces postes varie donc au gré des priorités du moment. coordinateur de la task-force interministérielle Ebola a été créé en novembre 2014 et supprimé à la fin de 2015 ; un ambassadeur thématique chargé de la présidence française du G7 a été nommé en janvier 2018, jusqu'à la fin de l'année le représentant spécial pour le numérique s'est vu reconnaître le statut d'ambassadeur thématique en 2018, compte tenu de l'ampleur prise par cette problématique ; les conférences Pékin+25 et le sommet Afrique-France organisés en 2020 ont conduit eux aussi à la création de postes d'ambassadeurs thématiques. Sur ces 21 postes relevés cette année, deux ne sont pas rémunérés,

nous faisons appel à telle ou telle personnalité pour assurer cette responsabilité. Tout cela est d'une grande clarté. La nomination se fait en conseil des ministres et, quand la mission est terminée, le poste

M. Olivier Cadic. Cet amendement a pour objet le dispositif « Français langue maternelle » (FLAM), qui vise à soutenir des associations proposant à des enfants français établis à l'étranger, dans un contexte extrascolaire, des activités permettant de conserver la pratique du français en tant que langue maternelle et le contact avec les cultures française et francophones. Les associations peuvent ainsi bénéficier de subventions d'appui au fonctionnement au démarrage de leur projet, ainsi que pour l'organisation de regroupements régionaux d'associations FLAM. L'opérateur désigné par le MEAE pour la gestion administrative du dispositif FLAM est l'AEFE. Cet amendement vise à la fois à développer le programme FLAM, en lui affectant un budget dédié, et à en transférer la gestion à l'Institut français, dont la mission est justement d'assurer la promotion de la langue française en s'appuyant sur un réseau d'alliances françaises et d'instituts bien plus développé et décentralisé que celui de l'AEFE, ce qui permettrait de toucher davantage de familles.

toute la jeunesse française expatriée puisse bénéficier d'un enseignement du français, de différentes façons. Pour autant, je ne suis pas favorable à cet amendement, parce qu'on ne peut déshabiller Pierre pour habiller Jacques. S'il faut octroyer des moyens supplémentaires au réseau FLAM,

qui sont une vraie réussite et des acteurs très importants pour nos compatriotes à l'étranger qui n'envoient pas leurs enfants dans les écoles françaises. Cela me paraît peu judicieux pour des raisons éminemment pédagogiques.

25 %, pour un montant total de 6,5 millions d'euros. Les recettes sont en effet en progression, et il nous a semblé que

Monsieur le ministre, vous nous avez expliqué que les ambassadeurs thématiques non diplomates effectuent un travail formidable et que tout va très bien.